J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux outre-mer a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable demande que le délai limite de dépôt des amendements de séance sur le projet de loi d'orientation des mobilités examiné en nouvelle lecture soit reporté du mercredi 30 octobre au lundi 4 novembre à douze heures. Y a-t-il des observations ?

Dans la discussion générale, la parole est à Jean-Marie Bockel, auteur de la proposition de résolution.

du président Gérard Larcher et conformément à notre mission de simplification des normes applicables aux collectivités, prend sa part de cet effort. Je citerai,

Pour autant, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Il faut rappeler quelques chiffres qui illustrent la difficulté de réduire significativement le flux des nouvelles normes et le stock des anciennes. Pour le flux, chaque année, sont publiés environ 50 à 60 lois, hors conventions, entre 1 600 et 1 800 décrets, près de 8 000 arrêtés ministériels et entre 1 300 et 1 400 circulaires. Quant au stock, il s'établit à plus de 80 000 articles législatifs et plus de 240 000 articles réglementaires en vigueur. en vigueur. Confrontés à cette difficulté, les pouvoirs publics se sont tournés vers une nouvelle méthode. Elle consiste à réduire le poids des normes en aval de leur production, d'une part, en sollicitant des services de l'État une interprétation « facilitatrice » de ces normes, d'autre part, en confiant à certains préfets, dans le cadre d'une expérimentation, le pouvoir de déroger à quelques-unes d'entre elles. Si nombre de préfets font de l'interprétation facilitatrice des normes, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire naturellement, il n'en reste pas moins que cette méthode est difficile à évaluer. Fondée sur de simples et lapidaires circulaires, elle ne dispose que d'une base juridique fragile et n'a fait l'objet d'aucun suivi par l'administration. Le pouvoir de dérogation aux normes s'appuie, quant à lui, sur une base juridique autrement plus solide : un décret de décembre 2017. Expérimenté depuis le mois d'avril 2018 dans vingt départements et régions, il permet aux préfets, dans un nombre limité de domaines, de déroger aux seules décisions individuelles relevant de leur compétence et fondées sur des mesures réglementaires. Nous avons pu évaluer ce dispositif, qui fait l'objet d'un véritable suivi par le ministère de l'intérieur. Et nous avons constaté qu'il joue d'ores et déjà un rôle utile dans les territoires où il est expérimenté.

nous semble donc devoir être pérennisé, étendu à tout le territoire, avec un champ d'application élargi. C'est l'objet principal de cette proposition de résolution, déposée par Mathieu Darnaud, aujourd'hui excusé, mais partie prenante de la démarche, et moi-même, que d'encourager le Gouvernement à le faire rapidement. je souhaite commencer par rappeler un point de méthode. Il est regrettable que, faute de suivi, l'incidence des instructions relatives à l'interprétation facilitatrice des normes soit impossible à mesurer.

par le ministère privilégie un dialogue direct avec les préfets expérimentateurs, chevilles ouvrières du dispositif. Elle pourrait par ailleurs associer des élus, des professionnels du droit, de même que le Conseil national d'évaluation des normes applicables

Une instance similaire avait été proposée par Alain Lambert et le regretté Jean-Claude Boulard, de même que par les rapporteurs de notre délégation, François Calvet et Marc Daunis, pour remédier aux difficultés du dialogue entre collectivités et services de l'État, en particulier pour ce qui concerne les projets d'urbanisme. Loin d'être une instance de plus, cette conférence départementale est une occasion de blocage et d'incompréhension. Au-delà de ses compétences inscrites dans la loi- l'émission d'un avis sur des cas complexes d'interprétation des normes ou sur les dérogations sollicitées -, elle serait par ailleurs un aiguillon pour les préfets et pour les services de l'État. J'ai bon espoir que cette instance finisse par voir le jour.

La recherche de la souplesse dans l'application du droit et l'objectif de simplification normative doivent devenir des éléments de la culture professionnelle des agents publics, pour l'instant davantage fondée sur le strict respect de la règle. Cela ne sera possible qu'en transformant les cursus de formation. Il est indispensable d'inclure des modules de formation initiale et permanente contre l'inflation normative dans les programmes des écoles du service public, les instituts régionaux d'administration, les IRA, Les témoignages des élus et des fonctionnaires territoriaux attestent, par ailleurs, de l'existence d'un déficit d'information sur les dispositifs de simplification qu'il est impératif de combler. À titre d'exemple, les sites internet des préfectures et du ministère de l'intérieur devraient comporter des rubriques aisément accessibles sur ces sujets. Cela étant, l'expérience montre que mettre en oeuvre la dérogation exige un surcroît d'instructions pour les services. Dans ces conditions, que l'administration centrale tienne compte de la dynamique facilitatrice des préfectures dans l'affectation de leurs moyens humains pourrait être non seulement une exigence de bonne administration, mais aussi un outil de motivation des personnels et des préfets. Enfin, quatrième et dernier axe, nous proposons d'élargir le champ de la possibilité de déroger aux normes. Il s'agit, d'abord, de l'ouvrir à l'ensemble du territoire national. Au-delà, une première faculté d'extension du champ d'application du décret consisterait à élargir la dérogation à des domaines nouveaux. Les préfets pourraient ainsi déroger en toutes matières relevant de leurs compétences, sous les réserves classiques du respect des engagements de la France et des intérêts de la défense ou de la sécurité. Par ailleurs, les « circonstances locales conditionnant la possibilité d'une dérogation préfectorale sont superfétatoires avec la condition de l'existence d'un motif d'intérêt général et ne semblent pas constituer une condition indispensable.

un puissant outil de déconcentration, consisterait à donner la faculté au préfet de département, selon des modalités à préciser, de déroger à des décisions relevant de la compétence des autorités supérieures, préfet de région ou ministre. Une troisième avancée, plus audacieuse, serait d'attribuer, cette fois aux autorités décentralisées, un pouvoir de dérogation sur les actes individuels relevant de leurs compétences. Une quatrième piste, plus ambitieuse encore, consisterait à autoriser des dérogations, sollicitées par les collectivités territoriales, à des normes législatives ou réglementaires.

N'oublions pas que pour les partenaires des collectivités et pour les citoyens, la différenciation territoriale peut être une source d'insécurité juridique et de complexité. Il lui faut donc un cadre d'exercice minutieusement construit,

certainement d'une intention louable : pérenniser les dispositions du décret du 29 décembre 2017, qui met en place l'expérimentation, sur quelques territoires choisis, d'un droit de dérogation des préfets à adapter la réglementation aux situations locales. Elle entend aussi, avant même de disposer d'un corpus suffisant de résultats de l'expérimentation en cours, élargir le domaine de cette expérimentation et populariser les exemples de dérogations réussies au titre de bonnes pratiques, ce qui nous paraît, cette fois, plus discutable. Je résumerai simplement mon propos. Premier point, le décret lançant l'expérimentation de ce droit préfectoral à déroger aux normes réglementaires est bienvenu et d'ailleurs étonnamment clair,

une adaptation de la réglementation serait souhaitable, cette instance ne saurait être, selon nous, transformée en instance d'expertise et encore moins en instance de décision,

il faut être moderne ! En outre, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on dit, les bonnes pratiques sont rarement généralisables réussite suppose le plus souvent des conditions locales très particulières. En faire la publicité avant une expérimentation suffisamment large me semble donc un peu risqué. je crains que tout l'appareil prévu par la proposition de résolution afin d'affermir juridiquement les décisions dérogatoires prises pour sécuriser les préfets et les inciter ainsi à se saisir de ce nouveau droit n'ait l'effet inverse : refroidir toutes leurs velléités d'innovation.

du poids des normes en aval de leur production, sorte de cauchemar récurrent de l'ensemble des élus locaux. La réduction du nombre de normes est évidemment une préoccupation extrêmement importante, régulièrement exprimée au Sénat. On le sait, un peu plus de 400 000 normes réglementaires s'imposent aux seules collectivités locales et les enferment très souvent dans un coûteux carcan juridique. Cette « incontinence normative », pour reprendre les termes employés par MM. Lambert et Boulard dans leur rapport de 2013, est un obstacle considérable à l'initiative. Elle est surtout contreproductive à l'efficacité de l'action publique, qui nous est chère et dont nous n'avons cessé de parler pendant ces quinze derniers jours. Elle l'est dans un contexte de crise économique et de baisse des ressources des collectivités. Les normes sont souvent, nous n'arrêtons pas de le dire, un empêchement de faire ! Mais ce matin, nous débattons plus spécifiquement du pouvoir de dérogation aux normes attribué aux préfets, une sorte de rêve pour les élus locaux, qui constitue un aspect important de cette thématique. Il convient en effet de s'intéresser aux outils qui permettent d'accompagner avec souplesse et pragmatisme les élus sur le terrain, à savoir l'« interprétation facilitatrice » et le pouvoir de dérogation des préfets. Et ce que nous examinons ce jour est bien, mes chers collègues, une facette de la différenciation territoriale. On ne cesse de parler de différenciation territoriale depuis plusieurs mois, à commencer par le Gouvernement. Ce fut en effet un axe très important du dernier discours de politique générale du Premier ministre, et Mme la ministre Jacqueline Gourault

Aujourd'hui, il est question d'une forme particulière de différenciation, qui concerne non pas l'organisation territoriale, mais l'adaptation des normes ou, plus précisément, l'adaptation des normes à la diversité et à la spécificité des territoires. Rappelons-le très très fortement, différenciation rime avec déconcentration. Il n'y aura pas de différenciation sans déconcentration

de déroger à des décisions relevant de la compétence des autorités supérieures » : il faut que les préfets aient cette possibilité de dérogation. C'est une nécessité pour commencer à s'extraire de l'inertie de la technostructure administrative à laquelle il arrive d'être un peu trop conceptuelle et normative.

cette deuxième proposition est liée à la précédente. Là encore, la finalité est que les élus aient face à eux une autorité pleinement déconcentrée et sécurisée, une autorité qui représente l'État, mais à laquelle on a conféré

de déroger, sur leur demande, aux normes législatives ou réglementaires relatives à leurs compétences, sous réserve d'un mécanisme politique empêchant la survenance d'abus et garantissant et garantissant l'égalité des citoyens devant la loi » : cette dernière proposition, probablement la plus ambitieuse, serait une nouvelle étape fondamentale de la décentralisation. Une décentralisation qui ferait le choix de la différenciation, d'une adaptation aux réalités locales avec, comme priorité, l'amélioration de la qualité des politiques publiques au bénéfice de nos concitoyens. Si nous appelons de nos voeux ces évolutions, je partage pour autant

qui, une fois installés, seraient difficiles à corriger. » Je tiens à saluer, une fois encore, la qualité du travail de nos deux collègues, Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud. Nous espérons que leurs propositions seront entendues par le Gouvernement dans les mois à venir, notamment dans le cadre du projet de loi 3D.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais féliciter M. le président de la délégation aux collectivités territoriales, Jean-Marie Bockel, et Mathieu Darnaud pour la proposition de résolution que nous examinons ce matin.

Prolifération », « inflation », « surproduction », les dénominations sont nombreuses pour désigner un mal désormais bien identifié : l'accumulation des normes qui pèsent sur les collectivités territoriales. On fait souvent remonter la prise de conscience de la prolifération des normes au rapport public du Conseil d'État de 1991, lequel établissait le constat suivant la surproduction normative, l'inflation des prescriptions et des règles ne sont pas des chimères mais une réalité ». De substantiels développements venaient étayer la démonstration de l'existence d'une véritable « logorrhée législative et réglementaire le constat est le même et se révèle particulièrement préoccupant pour les collectivités territoriales. À la demande du président Gérard Larcher et en emboitant le pas de Rémy Pointereau,

adoptée à l'unanimité par l'ensemble des groupes du Sénat en 2016. Nous avions, en effet, constaté les difficultés du dialogue entre collectivités territoriales et services de l'État, en particulier pour les projets d'urbanisme et d'aménagement. Une application stricte du contrôle de légalité n'est-elle pas un facteur d'absence de possibilité de dérogation ou d'adaptation nécessaire à la réalisation d'un projet de développement économique et créateur d'emplois ?

que cette idée d'une instance de conseil auprès du préfet n'ait, pour le moment, pas été suivie d'effet, alors même que constats de terrain et études montrent que les relations entre collectivités et services de l'État se sont dégradées depuis plusieurs années.

Je veux aussi évoquer deux points qui ne figurent pas dans la proposition de résolution. Le premier concerne plus particulièrement les zones frontalières où les transpositions de directives européennes ont ajouté des normes qui créent des distorsions de concurrence pour nos entreprises frontalières.

qui permettrait non seulement de corriger l'application des normes, mais également d'anticiper leur incidence sur le terrain. On ne peut plus se contenter des études d'impact du seul Gouvernement qui sont souvent insuffisantes, légères et, comme l'a souligné notre collègue Jean-Marie Bockel, orientées. Enfin, il s'agit non de dérogation aux normes, mais de différenciation. Comme l'a évoqué Mathieu Darnaud, la différenciation prend en compte une certaine dynamique territoriale suffisamment spécifique, comme en zone de montagne. On doit permettre de sortir du champ national. Ce texte pragmatique constitue un outil indispensable au service de la simplification du droit dans les collectivités territoriales. Il prend toute sa place dans la démarche d'ensemble suivie aujourd'hui pour lutter contre la surproduction des normes. est le sens des travaux menés au Sénat. En effet, s'il est vrai que de nombreux rapports ont permis d'affiner le constat, il n'empêche que les normes se multiplient, créent la complexité et induisent des coûts au détriment de l'efficacité de l'action publique.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il suffit de fréquenter les associations d'élus et d'assister à des réunions de maires pour se rendre compte que le thème des normes est omniprésent : « trop de normes Il faut regarder cela avec une certaine philosophie, car les mêmes qui protestent l'après-midi contre l'abondance des normes sont susceptibles d'en d'en demander davantage le matin, dans un juste souci de préservation de l'environnement, de sécurité ou de santé publique. C'est vrai ! Cela étant dit, il est vrai que la question se pose. Comment y répondre ? Cher Jean-Marie Bockel, cher Mathieu Darnaud, nous ne sommes pas persuadés que la solution passe par les préfets et leur pouvoir d'adaptation.

tout projet de texte réglementaire ou législatif susceptible d'entraîner des normes complémentaires pour les collectivités

éprouve des difficultés à formuler un avis dans les délais qui lui sont impartis. Il me semble qu'une des pistes serait de lui donner plus de moyens

sujets. Venons-en à nos préfets. J'ai une idée, peut-être simpliste- mais je ne crois pas -, de la fonction de préfet.

d'un État arbitraire prenant des décisions différentes en fonction des demandeurs et des collectivités territoriales concernées. » C'est ce que dit un préfet de la République ! Je fais également que M. le préfet de Vendée a utilisé cette possibilité d'expérimentation des dérogations dans une décision en faveur d'un parc éolien en évitant la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique.

résolution, parce que nous sommes attachés à la distinction des rôles et à la séparation des pouvoirs. La décentralisation n'est pas la négation de l'État

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que la réforme constitutionnelle, qui doit consacrer le droit à la différenciation territoriale, peine à voir le jour, le Sénat est réuni ce matin pour affirmer sa position sur le pouvoir de dérogation aux normes attribué aux préfets. Dans un pays historiquement centralisé tel que le nôtre, les normes ont toujours été conçues pour garantir une égalité de traitement entre les citoyens et les territoires, avec de surcroît des attentes très élevées envers les politiques publiques. Le constat est connu, ancien et unanime : chacun déplore l'inflation normative, législative comme réglementaire.

Le groupe RDSE y a pris sa part, avec le rapport de notre collègue Nathalie Delattre. La présente proposition de résolution constitue une nouvelle pierre à cet édifice titanesque. Mon groupe valide bien entendu sans réserve le rapport sur lequel elle s'appuie. Par son attachement aux territoires et à leur diversité, comme vous tous, il souscrit pleinement à l'objectif d'allégement des démarches administratives et d'accélération des procédures. Au-delà de la différenciation territoriale, le Gouvernement a reconnu que la réduction du stock des normes applicables aux collectivités figurait parmi les enseignements du grand débat. Ce n'est pas nouveau. Je pense aussi au travail important fourni par nos anciens collègues Alain Lambert et Jean-Claude Boulard dans leur rapport. Les élus nous le disent tous les jours : le poids des normes et des obligations alourdit leur charge de travail et ralentit la progression des réformes. L'inflation normative- je parle ici des flux, et non du stock -est un obstacle aux initiatives locales. Elle paralyse l'action publique, là où nos concitoyens attendent beaucoup des collectivités. Et elle alimente encore la crise des vocations chez les élus locaux. Bien entendu, les gouvernements successifs ont tenté ces dernières années de maîtriser cette inflation normative en réduisant non pas le flux de nouvelles normes ou le stock de normes anciennes, mais le poids des normes, grâce à une interprétation facilitatrice de la part de l'État et à une expérimentation offrant un pouvoir de dérogation aux préfets. L'interprétation facilitatrice étant soumise à un engagement concret des préfets, les auteurs de la proposition de résolution lui préfèrent le pouvoir de dérogation aux normes, qui s'appuie sur une base juridique plus solide et plus objective. Toutefois, cette expérimentation n'est pas exploitée à son maximum, puisqu'elle est mal connue et très encadrée. De plus, nous l'avons compris, elle arrive à son terme au mois de décembre prochain.

La différenciation territoriale pouvant être source d'insécurité juridique et de complexité, elle doit en effet être encadrée, pour être mieux conciliée avec le principe d'égalité des territoires. Toutefois, avant toute révision constitutionnelle, le groupe RDSE se joint à la délégation aux collectivités territoriales pour solliciter de l'État un indispensable desserrement des contraintes pesant sur les collectivités. Comment pourraient agir efficacement les petites collectivités face aux 1 600 décrets et 8 000 arrêtés ministériels produits chaque année alors que le contrôle de légalité des préfectures est de moins en moins protecteur ? la décentralisation propose ainsi plusieurs mesures pour davantage de rapidité, de souplesse et de pragmatisme dans la mise en oeuvre des politiques publiques d'abord, en rendant pérenne et en élargissant le champ d'application du droit à la dérogation pour les préfets de région ; ensuite, en donnant la possibilité au préfet de département de déroger à certaines décisions du préfet de région et du ministre enfin, en étendant également ce pouvoir aux collectivités qui souhaiteraient déroger à certaines normes pour tenir compte de leurs spécificités locales. Ces mesures seraient utilement complétées par une meilleure information des agents, élus et destinataires des normes, un dialogue local renforcé entre l'État et les collectivités, ainsi que par une meilleure évaluation du dispositif. Une consultation du Sénat est même envisagée pour les dérogations sollicitées par les collectivités. Assorties de telles garanties, les mesures évoquées semblent répondre au besoin de simplification de nos territoires. C'est pourquoi le groupe RDSE votera majoritairement en faveur de cette proposition de résolution. Toutefois, nous nous accordons pour dire qu'une démarche au cas par cas est limitée. C'est une approche globale dont nous avons besoin, pour ouvrir une nouvelle forme de décentralisation et de proximité. Cela passe par une profonde transformation des processus de fabrication des normes, au-delà de la seule révision constitutionnelle. Enfin, je tiens à rappeler que la dérogation doit poursuivre un motif d'intérêt général et de non-régression. Ne tombons pas dans la caricature en allégeant tout et partout. Le niveau d'exigence doit absolument être maintenu, notamment en matière environnementale, où l'idée de bien commun doit toujours nous accompagner. La parole

Nous sommes là pour nous livrer à une analyse du résultat produit par deux circulaires et un décret qui s'étalent entre 2013 et 2017, les circulaires parlant de « marge d'interprétation et le décret parlant, comme c'est logique, de « pouvoir de dérogation encadré ». Je participe à la demande générale de restitution et d'évaluation

donc de faire revenir dans l'application du droit une marge de pouvoir discrétionnaire. Simplement, le pouvoir d'appréciation se heurte à une peur et à une méfiance,

La rigidité de la loi ne vient pas de nulle part. Toute norme exigeante a été exigée. Dans le dialogue que nous avons avec la « société civile », selon le terme gramscien par lequel on a choisi de la baptiser, nous faisons en permanence face à des injonctions, à des demandes de règles fixes et transcendantes, à une démarche souvent très péremptoire ; et, disons-le, nous y cédons souvent.

très rigides, des lois que nous appliquons, la part de transpositions de textes de l'Union européenne est dominante.

de la rigidité de la loi et de l'exigence des procédures. Si vous êtes un bon avocat en matière d'environnement, vous gagnez tous vos procès sur des questions de procédure, jamais sur une question de fond. D'ailleurs, pour trouver une norme de fond dans le code de l'environnement, que j'ai un peu fréquenté, il faut se promener longtemps Nous sommes donc face à un enjeu qui touche très profondément la culture juridique de ce pays. Si nous voulons aller plus loin dans la transformation de méthodes de l'action publique, nous devons effectuer un travail de formation permanente de révision des concepts auprès de l'ensemble des services juridiques de nos services publics, ce qui est une vaste mission. Dans la vie de la plupart de nos institutions, on demande au service juridique de la sécurité. de la sécurité. Sa préoccupation va donc être de multiplier les précautions dans le sens du respect toujours le plus prudent, le plus scrupuleux, des règles de procédure en vigueur.

80 %, et je suis modeste, du pouvoir d'appréciation des autorités de commandes publiques est effacé par la préoccupation de sécurité inspirée par le service, dont c'est pour l'instant la conception de sa mission. Nous avons donc devant nous, me semble-t-il,

attribué aux préfets, déposée par nos collègues Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, deux spécialistes de la vraie vie des territoires. Ce texte s'inscrit dans la continuité des travaux menés depuis plusieurs années par notre institution, au service de la simplification du droit applicable aux collectivités.

celui des difficultés qu'ont les gouvernements successifs à y faire face, alors qu'un « choc de simplification » avait pourtant été promis voilà plusieurs années, mais en vain. Le résultat de cet état de fait est un environnement normatif encore trop souvent résistant à l'initiative locale, quand il ne lui est pas activement hostile. Face à cela, nos collègues invoquaient la nécessité d'un nouveau modèle, fondé sur le dialogue de l'administration centrale avec les échelons locaux. Je me joins à ce voeu, dont la réalisation s'impose plus que jamais, alors que, partout en France, de plus en plus d'élus locaux nous font connaître leur découragement. dans ce contexte qu'intervient la proposition de résolution dont nous discutons aujourd'hui. Elle traduit l'une des principales propositions du rapport : la possibilité pour les représentants de l'État de se faire les chevilles ouvrières d'une simplification flexible flexible et locale par le recours renforcé à des pouvoirs de dérogation aux normes. En réalité, des préfets remplissent déjà ce rôle. Depuis un décret du 29 décembre 2017, ils peuvent déroger L'expérience a été concluante. Dans certains cas, elle a permis d'économiser beaucoup de temps ou d'argent, voire de « sauver » des dossiers de subventions apparemment condamnés à échouer. Il est donc proposé, très justement, dans le présent texte d'étendre et de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif. aussi suggéré de développer les mécanismes de concertation entre services de l'État dans les territoires et les collectivités, et de mettre en place un meilleur suivi des résultats de ces mesures. Je pense qu'affiner les retours en provenance du terrain ne peut être que positif, aussi bien pour les collectivités que pour leurs partenaires au sein des directions locales de l'État. J'espère que le Gouvernement entendra cet appel à la coopération locale.

et ouvrir des possibilités de dérogation ne sert à rien si personne n'est averti de l'existence de celles-ci. C'est pour cela que rassembler les bonnes pratiques au sein d'un guide diffusé aux préfectures et communiquer sur ces problématiques est indéniablement une bonne idée. En plus, la mise en oeuvre en serait aisée et relativement peu onéreuse. cette proposition de résolution n'est évidemment pas une panacée. Il permet néanmoins d'ajuster le curseur de certaines situations sur le terrain et donc de mettre un terme à des symptômes. Mais nous ne devons pas cesser de nous efforcer de combattre le mal,

cette semaine, a été un signal fort quant aux souhaits d'évolution. La chambre des territoires est particulièrement attentive à la situation des collectivités locales, qui sont touchées par la multiplication des règles, l'inflation législative et la complexification des normes,

de l'accessibilité peut, pour des questions financières, mettre en difficulté une petite commune. Elle a également des répercussions sur nos hôtels et restaurants de campagne pour lesquels il est complexe, au regard de la faible rentabilité, de se mettre en totale conformité avec l'ensemble de la réglementation.

personnes handicapées pour l'arbitre, ou encore dans le secteur agricole. Sans la mise en place de normes très contraignantes, des subventions peuvent être refusées aux collectivités. L'expérimentation prévue par le décret du mois de décembre 2017 fut un exercice riche d'enseignements. Ce pouvoir utilisé environ une soixantaine de fois a montré que l'adaptation aux territoires était une nécessité rendant plus efficace l'application de la loi. Le lien entre l'échelon local et l'échelon national doit continuer à se construire et cela passera par un lien plus fort entre les services de l'État et les collectivités territoriales. L'écoute des élus locaux est primordiale, notamment celle du maire, qui connaît son territoire et les besoins de ses administrés. Sur ce point, la création d'une instance départementale permettant d'interpréter la norme la norme ou d'identifier les difficultés dans la mise en oeuvre de la norme à l'échelle locale nous paraît essentielle. La création d'un guide de bonnes pratiques et d'un processus d'information est tout aussi importante. Elle permettra une fluidification dans les échanges. La mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation est également nécessaire. La pratique nous démontre que nous devons constamment veiller à ce que la réglementation reste adaptée aux spécificités locales. une et indivisible, mais ses territoires ne sont pas les mêmes. Cela constitue sans doute notre richesse, mais rend parfois contreproductive une administration trop centralisée, chaque territoire présentant des spécificités et des handicaps Il nous faut identifier le problème avec précision. Il me semble qu'il est double : inflation normative et inadaptation aux territoires. le pouvoir de dérogation des préfets, à l'écoute des maires et des acteurs du territoire, va dans le bon sens. Mon groupe est convaincu qu'une plus grande décentralisation pourrait régler nombre de difficultés évoquées précédemment. De plus, nous devrons mener des discussions sur les matières auxquelles ces dérogations pourront s'appliquer, ainsi que sur les objectifs et les conditions de celles-ci. Ce travail préalable est nécessaire et nous permettra d'offrir un cadre précis et une définition claire de la consolidation du pouvoir de dérogation. mes chers collègues, oui à l'adaptation des normes aux territoires, oui à la simplification et à la souplesse normative, oui à la décision d'adapter la loi en fonction des territoires et des collectivités.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis le début du mandat, le Gouvernement partage une conviction : il faut répondre aux questions des territoires en fonction des territoires. Notre République est une et et indivisible, et je suis naturellement profondément attaché à ce principe de notre Constitution. Toutefois, l'unité signifie que nous devons trouver les meilleures manières de faire appliquer nos lois, les meilleurs moyens de faire valoir les principes de la République. Nous ne pouvons donc pas être aveugles face aux problématiques différentes des territoires et qui appellent, pour une même fin, des moyens parfois distincts.

qui permet une gestion au cas par cas plus efficace et pragmatique de certaines questions clés, comme l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'emploi et l'activité économique, ou encore la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel. Nous avons mis certaines contraintes et conditions à cette expérimentation. Ainsi, celle-ci doit être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales- j'y reviendrai. avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. Elle doit encore se limiter à la dérogation à des normes de niveau réglementaire, à l'occasion de décisions individuelles. être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. Enfin, elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, pas plus qu'une atteinte disproportionnée aux objectifs fixés par les dispositions auxquelles il est dérogé. Cette expérimentation concerne un nombre limité de départements- dix-neuf -et court sur une période de deux ans. Cependant, dès maintenant, nous pouvons commencer à en saisir l'utilité et les bénéfices. De ce point de vue, je tiens à saluer le travail mené par la délégation aux collectivités

Je crois que, sur ce thème, nous avons tout intérêt à avancer ensemble et je constate par le biais de cette proposition de résolution des sénateurs Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud que nous regardons dans la même direction. La première vertu de cette proposition de résolution est qu'elle constate tout l'intérêt du pouvoir de dérogation aux normes des préfets. Sur ce point, le Gouvernement est en plein accord. Ensuite, ce texte Ensuite, ce texte comporte des avancées que je veux saluer. Je pense à la systématisation des mécanismes de suivi et d'évaluation. C'est une mesure saine, utile et profitable à tous. Je pense également à l'idée d'édicter un guide de bonnes pratiques, qui est particulièrement pertinent et pourrait servir à tous les préfets et aux collectivités. D'autres exemples me viennent à l'esprit, comme un effort de communication sur la simplification des normes. C'est une volonté que le Gouvernement partage, et je peux d'ores et déjà indiquer que plusieurs pistes sont étudiées, comme la création de contenus dédiés sur les sites gouvernementaux, des communications plus régulières auprès des membres du corps préfectoral, ou encore la création de modules de formation en la matière. en la matière. J'ajoute que certains des points soulevés dans la proposition de résolution sont déjà en partie mis en place. Je citerai à cet égard deux exemples. part, l'idée de consulter les préfets expérimentateurs, afin d'avoir un retour sur expérience, est évidemment judicieuse. Nous avons déjà engagé ce travail. Le texte propose également d'aller plus loin, notamment en associant les élus à cette évaluation. C'est une suggestion intéressante,

d'appel pour avis, au-delà de la consultation de leurs administrations centrales. En revanche, je ne vous cache pas une plus forte réserve sur l'idée de créer une instance départementale en matière de simplification. Comme je le disais à l'instant, il existe aujourd'hui d'ores et déjà des moyens faciles pour que les préfets bénéficient d'éclaircissements sur des points de droit précis ; il pourrait donc être redondant, voire un peu contradictoire, de créer cent commissions départementales sur la simplification administrative.

D'abord, il paraît important d'attendre le retour sur expérience et l'évaluation du dispositif avant d'en élargir le champ. Pour autant, il est clair que, dans son principe et pour les domaines où elle est pratiquée, cette expérimentation a permis de réelles avancées.

à des décisions individuelles. Il ne s'agit pas d'une différenciation territoriale qui consisterait à appliquer les normes différemment d'un territoire à l'autre. D'une manière générale, ces décisions sont prises

notamment avec des associations environnementales. Cet arrêté n'a pas été attaqué : c'est bien la démonstration de toute la pertinence de ce dispositif, qui fait appel à

! C'est justement pour cette raison que je ne partage pas l'idée de supprimer la notion de « circonstances locales » des conditions nécessaires pour déroger à une règle à une règle de droit général. Il me semble que nous créerions un champ d'application peut-être trop large ; or l'important aujourd'hui est bel et bien de mener une politique adaptée à chaque territoire. La notion de différenciation, défendue par le Gouvernement, s'inscrit pleinement dans cette logique. Aussi, il me paraît essentiel d'en maintenir la mention. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, cette proposition de résolution va dans le bon sens et répond à un besoin bien réel. Nous souhaitons de l'adaptation envers les territoires. Nous souhaitons une approche pragmatique et efficace. C'est pourquoi le Gouvernement est favorable au présent texte. Très bien discussion générale est close. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explications de vote. Je mets aux voix la proposition de résolution. Mes chers

La séance est suspendue.